Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que les auteurs de la demande disposent d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'inertie du système climatique mondial fait que l'histoire du climat des trente prochaines années est déjà écrite dans ses grandes lignes. S'il est indispensable que tous les pays, particulièrement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, prennent des mesures d'atténuation pour éviter un effondrement climatique dans la deuxième partie du siècle, ces mesures n'auront pas un effet immédiat sur les évolutions climatiques en cours. Toutes les prévisions montrent que nous n'éviterons pas, d'ici à 2050, un réchauffement global de l'ordre de 2 degrés par rapport à la période préindustrielle. La France doit donc se préparer à absorber un choc climatique inévitable. Le rapport que j'ai réalisé avec Ronan Dantec décrit ce que signifie concrètement un tel réchauffement pour notre pays, nos territoires et nos concitoyens. Nous y dressons la carte de France des dérèglements climatiques à venir et de leurs impacts, notamment en matière de risques naturels, de canicule, de sécheresse des sols ou de tensions sur les ressources hydriques. Nous identifions les défis économiques, sanitaires et sociétaux que la France, dans sa diversité territoriale, devra relever pour faire face à cette situation. Enfin, nous formulons dix-huit propositions pour donner un nouvel élan à nos politiques d'adaptation climatique, notamment au niveau des territoires, car c'est en grande partie à ce niveau que se jouera le succès de l'adaptation. Je voudrais, pour lancer le débat de notre assemblée autour de ce rapport, évoquer plus particulièrement trois enjeux. Le premier concerne l'adaptation du bâti et de l'urbanisme. Dans les outre-mer, le sujet central est l'évolution des normes de construction et des mécanismes d'assurance pour tenir compte d'un risque cyclonique qui va s'intensifier. Dans les zones soumises à un risque d'inondation ou de submersion, l'évolution des normes et des mécanismes assurantiels constitue également un objectif central. Mais c'est sur un troisième point que je voudrais surtout insister ici : l'adaptation du bâti à des vagues de chaleur plus intenses, plus longues et plus fréquentes. L'importance de cet enjeu a été soulignée par les deux canicules historiques de cet été. Il est particulièrement marqué en ville en raison du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Il va devenir plus aigu à cause du réchauffement, mais aussi du vieillissement de la population. Or, jusqu'à présent, ce sujet est resté assez largement absent des réflexions des professionnels et des pouvoirs publics. Nous proposons donc d'inscrire la question du confort thermique d'été au centre de la définition de la norme RT 2020. Cela peut être l'occasion d'engager l'évolution des représentations et des pratiques de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction. Notre réflexion doit également inclure la question des outils et des moyens financiers nécessaires pour soutenir la transformation du bâti, notamment à l'occasion des rénovations. Un deuxième enjeu majeur de l'adaptation concerne les politiques de l'eau. Il y a un consensus pour dire qu'elles doivent donner la priorité à une utilisation plus économe de la ressource, ainsi qu'aux solutions fondées sur la nature, telles que la désartificialisation des sols, la restauration des haies ou la préservation des zones humides. Nous n'y parviendrons pas sans faire évoluer les mécanismes de tarification de l'eau. C'est un chantier nécessaire, mais sensible. Cela ne se fera pas non plus sans préserver les moyens des agences de l'eau et, à ce sujet, j'attire l'attention du Gouvernement sur les dangers des mesures budgétaires de court terme. Par ailleurs, parce que les politiques de l'eau se définissent concrètement au niveau des bassins hydrographiques, il est indispensable de mobiliser plus activement tous les acteurs concernés localement pour faire émerger, sur cette question, des visions communes et des projets de territoire. Des exercices Des exercices de prospective, comme Garonne 2050, peuvent aider à enclencher ces dynamiques locales. Enfin, il faut oser poser la question du stockage. Pourrons-nous faire face partout aux besoins uniquement par des mesures d'économie de la ressource ou d'autres qui s'appuient sur la nature ? Je n'en suis pas sûr. Il ne faut donc pas exclure les solutions de stockage, mais plutôt soumettre chaque projet à une condition : faire la preuve qu'il est nécessaire et que sa réalisation ne se fait pas au détriment de solutions d'adaptation alternatives. Je terminerai par l'adaptation de l'agriculture. Ce secteur sera le plus perturbé par le changement climatique. Pour autant, nous ne devons pas adopter une position défensive et pessimiste. J'ai la conviction que l'agriculture constitue un atout dans la transition climatique. Elle n'est pas le problème, mais une partie de la solution, si elle engage les transformations nécessaires. En même temps, l'agriculture française est vulnérable ; elle est confrontée à une concurrence internationale féroce de pays qui ne respectent pas toujours des normes aussi exigeantes que celles qui lui sont imposées. Il n'y aura donc pas d'adaptation de notre agriculture, si nous ne soutenons pas les agriculteurs par un plan national d'adaptation. ainsi qu'il faut intégrer l'enjeu de l'irrigation de manière responsable, en développant le stockage de surface, là où il est nécessaire, mais en le conditionnant à des pratiques agricoles plus économes de l'eau et plus respectueuses de la biodiversité. Enfin, il faut faire évoluer les mécanismes de couverture assurantielle pour qu'ils deviennent un outil incitatif qui encourage les exploitants agricoles à réaliser les efforts d'adaptation nécessaires. La parole

en 2050 par rapport à l'ère préindustrielle. Notre rapport n'est ni catastrophiste ni fataliste ; il est néanmoins sévère sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques, au-delà de quelques grandes structures scientifiques qui, pour leur part, sont engagées dans la réflexion et produisent des préconisations précises. Il montre ainsi que les défis de l'adaptation au changement climatique ne sont pas insurmontables. Nous avançons dix-huit propositions pour la mener avec succès. Mon collègue Jean-Yves Roux a présenté plusieurs réponses sectorielles, concernant notamment l'agriculture ou le bâti. J'évoquerai pour ma part des leviers d'action plus transversaux. Le premier d'entre eux est une mobilisation plus large des territoires dans les politiques d'adaptation.

Mais vous n'ignorez pas, madame la ministre, le retard pris dans leur élaboration et leur adoption. Il est plus que temps de systématiser l'engagement des territoires au-delà des quelques collectivités pionnières, car c'est à cette échelle que se construisent les réponses pertinentes. Chaque territoire a en effet ses vulnérabilités particulières il a ses ressources propres et son projet de développement spécifique. L'adaptation ne peut donc pas être uniforme : elle se construit sur la base d'un diagnostic territorial précis, propose des réponses sur mesure et s'appuie sur un projet porté et partagé localement.

Il faut aussi conforter la fonction d'orientation stratégique des régions par la généralisation de prospectives régionales sur l'excellent modèle aquitain AcclimaTerra- on ne le citera jamais assez ! - ; ces prospectives portent un diagnostic précis des évolutions prévisibles à l'échelle de la région. Nous avons besoin de démonstrateurs régionaux et de contractualisation d'objectifs d'adaptation dans les financements régionaux. Le deuxième levier transversal de mobilisation sur lequel je veux insister est le soutien à la recherche et la simplification de l'accès aux données.

qui provoque l'incompréhension de la communauté scientifique. Or nous avons évidemment besoin d'évaluer tous les impacts du changement climatique sur la nature, la santé et l'économie et de comprendre les évolutions dans le temps, facteur clé des stratégies Nous avons donc besoin de connaissances pour nourrir notre action et nous avons surtout besoin que ces données soient rendues plus accessibles aux acteurs de terrain- c'est la clé de la mobilisation. Nous faisons pour cela plusieurs propositions : accentuer le soutien financier à la recherche et à l'expertise scientifiques ; accorder un accès gratuit, et surtout beaucoup plus facile, aux données nécessaires à l'élaboration des politiques d'adaptation territoriales, notamment aux scénarios de Météo France. Il y a, dans le Pnacc 2, l'idée d'un grand portail d'information de l'adaptation. Il doit associer l'ensemble des services et opérateurs compétents de l'État et être un véritable guichet unique d'un service public de l'adaptation- c'est une véritable priorité. troisième point essentiel concerne l'utilisation accrue du secteur assurantiel comme levier de transformation. Il faut s'engager dans une évolution des modalités de prise en charge par les assurances du coût des sinistres climatiques.

Je conclurai en évoquant une dernière proposition forte de notre rapport : un projet de loi-cadre sur l'adaptation de la France au changement climatique devrait être présenté au Parlement. pourrait être l'occasion d'inscrire enfin ce thème au coeur du débat public et d'en examiner de façon cohérente et transversale tous les aspects. Jean-Yves Roux a cité il y a quelques instants la question de l'eau. C'est un excellent exemple. Sur ce point, sans un compromis dynamique et une compréhension mutuelle entre acteurs, nous allons à l'affrontement- nous en et une compréhension mutuelle entre acteurs, nous allons à l'affrontement- nous en avons déjà de douloureux exemples. Cette loi doit fournir le cadre de cette concertation et donnera un signal fort sur le caractère prioritaire des politiques d'adaptation, en renforçant aussi, évidemment, la place du Parlement. La parole est

Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer la qualité de ce rapport qui dresse un constat sans appel, mais lucide, des impacts déjà observés en France et de

On peut les résumer ainsi : nous devons poursuivre avec acharnement la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, mais nous devons également nous préparer aux impacts que nos émissions passées rendent désormais inéluctables. Je souhaite vous présenter l'action conduite par le Gouvernement et l'accélération que j'ai l'intention de lui donner. La France est l'un des pays les plus avancés en matière de planification de l'adaptation : après une stratégie nationale en 2006, elle s'est dotée d'un premier plan d'action en 2011. En décembre 2018, le Gouvernement a publié le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, le Pnacc 2. Axe 19 du plan climat, il a pour objectif général de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour adapter la France dès 2050 à une hausse une hausse de la température moyenne de la Terre de 2 degrés par rapport à l'ère préindustrielle, en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris, mais à un horizon temporel plus proche de façon à ne pas exclure des scénarios de changement climatique plus pessimistes. Le Pnacc 2 comporte quatre priorités : la territorialisation de la politique d'adaptation, l'implication des filières économiques, le recours aux solutions fondées sur la nature et les outre-mer. cinquante-huit actions réparties en six domaines : gouvernance ; prévention et résilience ; nature et milieux ; filières économiques ; connaissance et information ; international. Les douze ministères concernés prévoient de consacrer 1,5 milliard d'euros sur cinq ans pour engager les actions de ce plan contre 171 millions d'euros pour le précédent, laquelle s'ajoutent les 500 millions d'euros par an que les agences de l'eau et leurs comités de bassin ont prévu d'investir à travers leur onzième programme d'intervention 2019-2024 dans des actions d'adaptation au changement climatique. Les leçons tirées du premier plan national d'adaptation au changement climatique nous ont montré qu'un suivi régulier du plan était nécessaire pour s'assurer de sa bonne mise en oeuvre par les nombreux acteurs impliqués. C'est pourquoi il fait l'objet d'une déclinaison opérationnelle avec un programme de travail annuel présenté à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, chargée de son suivi- elle est présidée par M. le sénateur Ronan Dantec. Le bilan Le bilan d'avancement du plan sera également présenté chaque année à la commission spécialisée et fera l'objet d'un avis du CNTE. Une série d'indicateurs de suivi est en cours en définition avec la commission spécialisée et une application informatique de suivi des actions a été développée par mes services et mise à la disposition des pilotes ministériels.

l'intégration du climat futur dans les modélisations de la stratégie nationale bas carbone ; le suivi de l'élaboration de trois normes internationales ISO sur l'adaptation au changement climatique ; le lancement

L'élaboration du Pnacc 2 ayant fait l'objet d'une concertation de deux ans avec près de trois cents représentants de la société civile, experts, représentants des collectivités territoriales et des ministères concernés, il est cohérent avec les dix-huit propositions de la délégation à la prospective du Sénat. On y retrouve notamment des actions relatives à l'éducation et la formation, ce qui rejoint la proposition 2 du Sénat, la volonté de synergie entre les actions d'atténuation et d'adaptation- proposition 3 le portage de cette problématique au niveau européen- proposition 4 -, la formation des élus- proposition 12 -, l'intégration du confort d'été dans les travaux sur la prochaine réglementation des bâtiments neufs- proposition 16 -et la question de la ressource en eau. Il me semble cependant que nous devons accélérer nos efforts. Les épisodes récents de canicule et de sécheresse ont rappelé que la France est d'ores et déjà exposée aux conséquences du changement climatique et que notre niveau de préparation à ces impacts doit encore être amélioré. Les territoires d'outre-mer sont particulièrement concernés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. La submersion marine peut y être aggravée par les cyclones. Le cyclone Irma a également mis en lumière les risques auxquels ces territoires sont exposés. C'est pourquoi je souhaite que le Pnacc 2 soit renforcé et que sa mise en oeuvre soit accélérée. Plusieurs actions nouvelles ou anticipées seront donc lancées. Je souhaite tout d'abord qu'un retour d'expérience exhaustif des deux épisodes de canicule de 2019 soit réalisé. soit réalisé. Il permettra de vérifier si le contexte législatif et réglementaire actuel est suffisant pour anticiper les impacts présents et à venir du changement climatique. Il permettra également d'analyser la façon dont le plan national canicule pourrait être étendu aux impacts autres que sanitaires selon les niveaux de vigilance de Météo France. La question du confort d'été devra également être intégrée dans le champ des réflexions en cours sur la rénovation des bâtiments publics.

La prévention des risques naturels est évidemment un enjeu crucial. Bientôt dix ans après la tempête Xynthia, nous ferons un point des nombreuses actions conduites et de ce qui doit être renforcé dans un contexte de hausse accrue du niveau des mers que le récent rapport du GIEC a bien mis en valeur la semaine dernière. Je veillerai à ce que les moyens requis, qui bénéficient en premier lieu aux collectivités locales, acteurs majeurs de la prévention des risques, soient préservés, accrus si besoin, et utilisés le plus efficacement possible au travers du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, Enfin, pour les territoires de montagnes, nous allons finaliser un plan de prévention des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Les suites du Livre bleu des outre-mer mettent en avant la question de l'encadrement des constructions pour diminuer la vulnérabilité aux cyclones. Je souhaite aussi que la résilience de nos systèmes de transports, déjà dotés de plans de continuité, entre autres, à la SNCF et à la RATP, soit renforcée au niveau des infrastructures, des matériels et de la gestion des pics de chaleur. Des actions sont conduites sur les réseaux électriques, tant pour les situations de forte chaleur que pour celles liées à des inondations. Un bilan sera utilement conduit pour voir si des accélérations sont nécessaires. Et nous avons bien d'autres idées ; je ne les citerai pas maintenant, mais je pourrai le faire durant notre débat. Je tiens à saluer la qualité du rapport présenté par MM. les sénateurs Dantec et Roux. C'est un sujet transversal qui concerne l'ensemble des ministères ; ils doivent naturellement mais le Gouvernement ne pourra pas à lui seul réussir l'adaptation de la France au changement climatique. Je souhaite une mobilisation de tous les acteurs. Le rôle des collectivités territoriales, que ce soit à travers les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou les plans climat-air-énergie territoriaux, doit être rappelé et soutenu. Il pourrait être utile de faire un point régulier sur ces aspects, par exemple en organisant un séminaire annuel à destination des collectivités locales et de leurs associations, ainsi que des parlementaires intéressés. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour réussir l'adaptation de notre pays au changement climatique. Nous allons

Ce week-end, j'étais invité à la pendaison de crémaillère d'un logement particulièrement intéressant : un bâtiment comportant plusieurs logis, intégré dans son environnement, économe en foncier, écologique et local. Ses matériaux sont issus du territoire : du bois de nos forêts, des blocs de chanvre pour les murs, de la terre issue des fondations pour les enduits et une toiture végétalisée intégrant des panneaux solaires et permettant la récupération d'eau. Ces matériaux biosourcés, trouvés sur place, peu chers, peu transformés, dont le bilan carbone est extrêmement faible, permettent de stocker des quantités de carbone considérables. Ces logements passifs, grâce à une isolation performante qui procure un confort thermique inégalable été comme hiver, ne nécessitent pas ou peu de chauffage. Cette maison respire, son hygrométrie lui permet de rafraîchir et d'assainir l'air ambiant. Pas besoin de système de ventilation gourmand en énergie ni de climatisation. Et si, demain, cette maison devait être démolie, elle retournerait là d'où elle vient, le sol ! Pas ou peu de déchets, puisque ces matériaux complètement biodégradables termineront leur cycle. Pour l'alimentation, nous utilisons l'expression « du champ à l'assiette », ici, ce serait plutôt « du champ au logis », avec la création de formes architecturales propres à chaque territoire, s'éloignant de l'uniformisation qui a déjà gommé les spécificités de nos régions. Ces habitations, madame la ministre, n'ont rien d'exceptionnel ; elles relèvent simplement du bon sens, principe qui est cher à cette assemblée. Et pourtant, ce type de construction est encore marginal. Il est nécessaire de lever les obstacles pour créer de véritables filières locales, faciliter la labélisation et la délivrance d'avis techniques pour ces matériaux, accompagner la mise en place d'une gestion durable de la ressource en bois, valoriser l'utilisation de la paille ou la culture du chanvre encore entravée par une réglementation absurde, ou encore adapter la formation des artisans en lien avec les besoins et les capacités de leur territoire plutôt qu'avec la standardisation des géants du BTP. Il s'agit d'une réponse concrète et d'une politique sociale et écologique, une politique qui peut être développée à l'échelon local

ainsi, 200 000 euros sont prévus dans le programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique. La construction en bois présente aussi de nombreux atouts : c'est un levier de développement économique des territoires ruraux et forestiers qui permet de stocker du carbone, ce qui constitue un levier important pour nos objectifs de neutralité carbone. C'est pourquoi la France s'est dotée, en 2017, d'un cadre stratégique pour l'ensemble de la filière au travers du programme national de la forêt et du bois qui précise les orientations stratégiques liées à la forêt et à et à l'ensemble de la filière bois. Les objectifs sont ambitieux : adapter les forêts au changement climatique, conserver le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et sécuriser en qualité, en quantité et en régularité La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments permettra de valoriser le stockage du carbone biogénique dans l'évaluation environnementale des bâtiments neufs. Je pense que nous pouvons encore progresser en la matière et nous devrons suivre avec attention la mise en oeuvre de ce programme.

Ronan Dantec et Jean-Yves Roux pour la qualité du travail qu'ils ont accompli avec la délégation à la prospective et pour l'ensemble des propositions qui sont présentées dans leur rapport.

des émissions antérieures sur des systèmes inertes comme les océans nous oblige tout de même à gérer un certain nombre de conséquences inéluctables pour le siècle actuel,

territoire, un certain nombre d'atolls sont appelés à disparaître. Nos outre-mer sont donc en première ligne sur ces questions d'adaptation au changement climatique,

la prospective, leurs travaux concernant les dérèglements climatiques. Les impacts du réchauffement sont ciblés, cartographiés selon les différentes régions de France, exposant clairement ce à quoi l'on peut s'attendre d'ici à 2050 et après. Considérant l'urgence et la nécessité du concours de chacun pour lutter contre les conséquences dramatiques du changement climatique, madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il faille créer une compétence « réchauffement climatique » dévolue à l'État, aux régions, aux départements, aux EPCI et aux communes, afin que chacun saisisse dès maintenant l'occasion d'anticiper et d'intégrer ces changements dans tout projet ? Par exemple, il faudrait permettre aux communes, à l'occasion de travaux ou de constructions, de prévoir des ouvrages de drainage ou de stockage d'eau, qui atténueront les inondations ou alimenteront les sites arides. Votre ministère peut, dès à présent, donner ses directives sans perdre des années dans l'élaboration d'un énième schéma régional. Certaines actions sont aussi simples qu'urgentes, et je crois qu'il serait judicieux de compter sur le bon sens local, celui des communes et des intercommunalités, notamment, pour mettre en place, au fur et à mesure de leurs réalisations, les moyens de lutter contre des fléaux parfois déjà installés. Encore faut-il leur en donner la compétence, les inciter et les accompagner financièrement dès à présent. La parole

passe par une mobilisation non seulement de l'État, mais aussi des régions et des intercommunalités. Précisément, la loi NOTRe a confié aux régions l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, un Sraddet, dans lequel doivent figurer les orientations sur l'adaptation au changement climatique. De leur côté, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un plan climat-air-énergie territorial, un PCAET, avec une série d'actions pour se préparer aux impacts du changement climatique. En tant que chefs de file climat-air-énergie, les régions ont naturellement vocation à animer, sur leur territoire, la thématique de l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, s'agissant des projets, ceux qui ont des impacts sur l'environnement doivent être accompagnés d'une évaluation environnementale et stratégique, puis faire l'objet d'une consultation du public avant d'être autorisés. Depuis 2016, cette évaluation doit, en particulier, analyser les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique. le climat et sa vulnérabilité au changement climatique. Ce diagnostic est nécessaire pour identifier et anticiper les fragilités des aménagements et de leurs usages. Cela permet ensuite de prévenir les dommages consécutifs au changement climatique sur les infrastructures

en conséquence, pour les travaux dans toutes les collectivités. Au-delà du soin apporté à la qualité des bâtiments, il faut se prémunir aujourd'hui des inondations, de l'assèchement, de la disparition de nos forêts, car les scolytes et autres parasites y font actuellement des ravages incommensurables. Il nous faut donc agir conjointement

l'équilibre urbain entre les quartiers, en réalité, très peu de textes sont extrêmement clairs et précis sur

qui ne me semble favorable ni au climat ni à la biodiversité ? Pour ma part, je suis convaincue qu'il faut, avec détermination, et

et l'érosion des côtes. Notre pays compte en effet de nombreux kilomètres de littoral. Aujourd'hui la densité de population est 2,4 fois plus élevée sur le littoral que la moyenne nationale et, d'ici à 2040, d'après l'Observatoire national de la mer et du littoral, 40 % de la population vivra sur les bords de mer. de la délégation, qui permet de donner une vision globale de l'ensemble des défis auxquels la France et le reste du monde devront faire face d'ici à quelques années, et qui nous donne également l'occasion d'interpeller le Gouvernement sur les risques climatiques et la gestion des catastrophes naturelles. En effet, avec les dérèglements climatiques, les catastrophes naturelles, qui sont souvent définies comme des épiphénomènes, vont devenir de plus en plus courantes dans les années à venir. Les Français et les élus locaux sont déjà, et seront de plus en plus confrontés aux dérèglements climatiques, et donc aux aléas climatiques comme les tempêtes, les sécheresses, les inondations, etc. Au vu de ces enjeux et de ces défis, il semble crucial de réorienter les politiques publiques dès maintenant et d'investir dans le service public pour protéger et accompagner les populations et les élus des territoires. et les élus des territoires. C'est pourquoi les dispositifs de prévention et d'accompagnement des élus locaux et des sinistrés doivent être placés à la hauteur des enjeux. Les changements climatiques entraînent des bouleversements profonds de nos écosystèmes au-delà des nécessaires évolutions de nos modes de vie ; ils bouleversent toute l'organisation de notre société. Madame la ministre, à quand des politiques ambitieuses, qui permettront d'accompagner ces changements en faisant les efforts nécessaires pour prévenir les conséquences du dérèglement ?

l'ensemble des conséquences, que l'on sait désormais inéluctables, de ce réchauffement climatique, que l'on peut d'ores et déjà constater.

proposées par le plan national d'adaptation au changement climatique sont tout aussi indispensables. Vous le savez, l'État agit pour accompagner nos concitoyens face à ces risques naturels qui peuvent s'aggraver.

qui est un outil majeur de financement de la politique de prévention des risques naturels. Il apporte en effet un soutien aux actions des collectivités locales.

Parmi ces dérèglements figure la survenue de vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus sévères. Nous en avons vécu deux successives cet été, qui ont aggravé une situation de sécheresse déjà bien présente depuis l'an dernier. Nos agriculteurs peuvent malheureusement en témoigner. Le rapport confirme ce que nous craignons tous : une augmentation de l'intensité, mais aussi de la durée, de la sécheresse des sols, qui passerait de deux mois actuellement, soit de mi-juillet à mi-septembre, à quatre mois d'ici à 2050, c'est-à-dire de mi-juin à mi-octobre. je parle ici de moyennes, puisque des restrictions d'eau sont encore imposées aujourd'hui dans bon nombre de départements. Le 21 août, le ministère de l'agriculture a autorisé l'exploitation des terres en jachère pour nourrir les bêtes, en raison de niveaux de stocks de fourrage particulièrement bas. Aujourd'hui, au-delà de ces mesures d'urgence, il est indispensable de penser et de mettre en oeuvre des solutions à long terme pour garantir la survie de l'agriculture française, qui est un modèle pour de nombreux pays. Parmi les idées qui émergent figurent les retenues d'eau, ou retenues collinaires. Ces structures sont destinées à recueillir l'eau de pluie et de ruissellement, notamment en automne et en hiver, pour la restituer à l'agriculture lorsque la pluie se fait plus rare. Une soixantaine de retenues devraient être autorisées par le ministère d'ici à 2022. Ma question est donc double pensez-vous que le stockage de l'eau soit la solution appropriée à encourager ? Plus largement, pensez-vous qu'en raison du changement climatique profond que nous vivons, il faudra, dans certaines régions, envisager une évolution globale des pratiques agricoles ? Très bien ! La parole

de réduire la vulnérabilité de l'agriculture à un risque accru de manque d'eau dans ce contexte. Vous le savez, le Gouvernement porte une attention particulière à la gestion durable de la ressource en eau. C'est tout le sens des travaux menés dans le cadre des Assises de l'eau, qui ont permis de donner les grandes orientations sur les politiques publiques relatives à la gestion de la ressource.

Les services de l'État sont mobilisés pour accompagner les territoires dans l'élaboration de projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE. Il est indispensable que toutes les solutions soient considérées. La recherche de sobriété et d'optimisation de l'utilisation de l'eau passe notamment par des réflexions sur des variétés mieux adaptées aux territoires, les solutions de stockage ou de transfert, et donc sur la transition agroécologique, qui est porteuse de solutions pour une meilleure résilience de l'agriculture face aux changements climatiques. Sur votre question très précise des retenues collinaires, je dirai que, d'une manière générale, le stockage artificiel de l'eau est une solution possible, parmi d'autres, pour répondre au problème du décalage dans le temps entre la disponibilité de l'eau et les besoins des cultures. Parmi les stockages artificiels,

voilà quelques semaines, les images de l'Amazonie en feu ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation internationale. Pour faire miennes des paroles si souvent prononcées ces derniers jours,

L'émotion passée, chacun s'interroge sur les conséquences terribles de ces incendies sur le climat. La première est évidemment la libération dans l'air d'une très grande quantité de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. C'est aussi la destruction de puits de carbone essentiels et de réserves de biodiversité exceptionnelles. La forêt amazonienne régule en partie, par son rôle fondamental dans le cycle hydrologique du bassin amazonien, le climat non seulement de l'Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. entier. L'assèchement provoqué par la déforestation et les feux dégrade enfin les cycles de l'eau et du climat. Selon certains scientifiques, la multiplication des grandes sécheresses exposerait l'Amazonie à un risque de « savanisation » qui, si elle advenait, tomberait comme un couperet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour être clair, on estime aujourd'hui qu'une déforestation de 20 % à 25 % de l'Amazonie pourrait faire basculer fatalement son climat. À ce jour, la forêt aurait déjà été détruite à plus de

est un enjeu majeur. Vous le savez, la France est un des premiers pays à s'être doté d'une stratégie nationale contre la déforestation importée.

le service « valorisation économique de la biodiversité », qui a récemment ouvert en Guyane, a vocation à apporter son appui pour, à la fois, permettre un développement de nos territoires et lutter contre la déforestation qui affecte encore trop souvent nos forêts équatoriales.

Le rapport Explore 2070 montre que la baisse de la recharge des nappes phréatiques est déjà amorcée. Deux territoires sont particulièrement affectés : le sud-ouest, dont mon département, le Lot-et-Garonne, fait partie,

Cette étude révèle aussi que, si des mesures immédiates ne sont pas prises, cela entraînera des conflits entre les différents usagers. Ainsi, tous les usages de l'eau, c'est-à-dire la consommation humaine, l'agriculture, le tourisme, la préservation des milieux aquatiques, seront affectés. est pourtant un pays d'abondance hydrique, grâce à son climat tempéré et à la multitude de ses fleuves et de ses montagnes. Pour améliorer le rapport entre les besoins et les ressources, on pourrait engager plusieurs actions simultanées inciter financièrement à la réduction de consommation d'eau ; partager la ressource entre les territoires où elle est plus ou moins abondante ; encourager le recyclage ; développer le stockage de l'eau en hiver avec la construction de nouvelles retenues collinaires et de haute montagne et le développement de nouvelles techniques de recharge des nappes phréatiques. Les sécheresses survenues pendant les étés de 2018 et de 2019 sont la démonstration que l'idéologie anti-irrigation, anti-stockage de l'eau

permettant de nourrir les populations et maintenir des étiages suffisants pour préserver la faune et la flore de nos fleuves, de nos rivières et de nos ruisseaux ? La parole est à Mme la ministre.

qui est le résultat des concertations et des travaux menés dans le cadre des Assises de l'eau, prévoit bien l'élaboration de projets de territoire pour la gestion de l'eau

eau potable, pour le maintien de la biodiversité, ce qui suppose un certain niveau d'étiage dans les cours d'eau, pour la lutte contre les incendies,

Du fait de son tissu urbain très dense, la ville génère un microclimat urbain dit « îlot de chaleur urbain »- mon collègue Roger Karoutchi en a parlé. Les augmentations de températures de 2 à 4 degrés prévues d'ici à 2050 et les canicules de plus en plus fréquentes seront donc encore plus difficiles à vivre pour les Parisiens. En outre, d'après une étude de septembre 2019 de, Paris est la ville française où l'isolation et la consommation énergétique des logements laissent le plus à désirer, avec une consommation annuelle moyenne d'énergie de 242 kilowattheures au mètre carré, soit une étiquette énergie E. En période de canicule, comme en période de vague de froid, la majorité des Parisiens peinent déjà à maintenir leur logement à une température décente, et je parle en connaissance de cause Les contraintes administratives, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique de copropriété, n'améliorent pas cette situation. En effet, seuls des travaux de rénovation énergétique pourront garantir aux Parisiens un confort d'été et d'hiver. Il est donc indispensable que l'État maintienne et intensifie les outils d'incitations. Je m'étonne donc de l'inscription dans le projet de loi de finances de la transformation du CITE en une prime attribuée en fonction des revenus des ménages. Ce nouveau dispositif ne va pas dans le sens de la lutte contre les passoires énergétiques et de l'objectif fixé par le Gouvernement, qui prévoit 500 000 rénovations énergétiques de logements par an. cette prime des ménages des deux derniers déciles de revenus- soit des foyers propriétaires plus enclins à réaliser les travaux que les locataires -et l'absence totale d'aide à la rénovation globale, pourtant la plus efficace, détourne cette réforme de son objectif initial. Madame la ministre, ma question est donc la suivante : comment le Gouvernement entend-il inciter les Français à adapter leur logement aux changements climatiques sans leur fournir des outils efficaces pour rénover énergétiquement leur habitation ?

Je souhaite donc connaître, madame la ministre, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour développer les PTGE, les fameux projets de territoire pour la gestion de l'eau,

départements ont pris des arrêtés de crise, imposant l'arrêt des prélèvements d'eau afin de préserver des usages prioritaires. L'adaptation au changement climatique nous demande de repenser les différentes composantes, de la prévention des sécheresses à la gestion de crise. Nous devons donc revoir, dans sa globalité, la gestion quantitative de l'eau afin de donner une place privilégiée aux solutions naturelles. Nous devons notamment désartificialiser des sols pour augmenter leur capacité d'infiltration et limiter le ruissellement. Nous devons préserver les milieux humides pour profiter de leur capacité de stockage. Nous devons restaurer des capacités de ralentissement des écoulements par des cours d'eau pour permettre aux espèces aquatiques de résister aux périodes de stress hydrique. Nous devons nous mettre en ordre de marche pour revenir à l'équilibre dans les bassins en déficit structurel d'eau. Tel est bien le sens de l'instruction

et des risques qu'elle entraîne sur la santé de nos concitoyens. Les risques liés à la pollution de l'air sont nombreux. Ils le sont en particulier pour les enfants en raison de l'immaturité de leur organisme et de la fréquence de leur respiration, plus élevée que chez l'adulte. C'est le cas de Timon, neuf ans, qui souffre depuis 2011 de bronchites et de toux liées à la pollution atmosphérique dans l'agglomération lyonnaise, fortement touchée par les concentrations en particules fines. Statuant sur une demande de réparation des parents de l'enfant, le tribunal administratif avait ainsi qualifié l'État de « fautif L'Unicef, qui rappelle que la principale source de pollution atmosphérique dans nos villes est le trafic automobile, fait état d'un chiffre plus qu'alarmant : trois enfants sur quatre respireraient un air pollué en France. Deux autres études montrent également que la pollution de l'air accroît le risque de mortalité infantile et réduit la fonction pulmonaire. Les enfants sont exposés à cette pollution au sein même des écoles de la République. En effet, la majorité des lieux d'accueil pour enfants se trouvant à proximité d'axes routiers, leur exposition à un air pollué est donc accentuée. Pourtant, des solutions existent soutenir les collectivités pour développer des réseaux de mobilités plus propres, à généraliser les zones à faibles émissions dans les villes ou encore à diminuer le trafic routier à proximité immédiate des établissements scolaires. Madame la ministre, face à l'urgence sanitaire, l'État a la responsabilité d'agir pour protéger les Français, les plus vulnérables en particulier. Aussi, pouvez-vous ici nous indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement mettra en oeuvre durant le quinquennat pour prévenir les risques sanitaires majeurs et sensibiliser la population ? La parole

métropoles ont répondu à l'appel que nous avons lancé à l'été 2018. Nous accompagnons désormais vingt-trois territoires sur lesquels vivent 17 millions de Français dans la mise en place de zones à faibles émissions.

de déployer des moyens de vidéoverbalisation, puis de contrôle-sanction automatiques, qui devraient se mettre en oeuvre respectivement à l'été 2020 et à l'été 2021. Je partage tout à fait votre préoccupation, qui est importante, même si elle n'est pas directement liée à l'adaptation au changement climatique. Nous devons agir place ces zones à faibles émissions. Il faut mettre en oeuvre une politique visant résolument à proposer des alternatives à l'usage de la voiture individuelle, dans nos métropoles, mais aussi sur le reste de notre territoire, là où nos concitoyens peuvent souffrir d'être dépendants de la voiture individuelle.

Celui-ci traite à plusieurs reprises des conséquences graves et rapides du changement climatique en zone de montagne. J'aimerais, à cet instant, revenir sur un enjeu majeur, qui aura un impact dépassant largement les zones de montagne. Il s'agit des débits d'eau. Il y a tout juste une semaine, le GIEC dévoilait son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Pour les glaciers, les prévisions sont alarmistes : 80 % de la surface des glaciers aura disparu en 2100 si les émissions continuent sur cette tendance. Or « tous les grands fleuves européens prennent leur source en montage ». Les Alpes assurent ainsi 34 % du débit moyen du Rhin, 40 % de celui du Rhône et 53 % de celui du Pô. D'ici à 2100, le réchauffement climatique devrait faire grossir les débits de ces fleuves de 20 % en hiver, les réduire de 17 % au printemps et jusqu'à 50 % en été. En d'autres termes, les populations vivant dans les plaines seront soumises à des risques accrus d'inondation en hiver et de sécheresse en été. Cela me conduit, madame la ministre, à vous alerter sur deux sujets d'actualité. Tout d'abord, la perspective d'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques nous fait redouter les conséquences sur la bonne maîtrise de gestion des crues et de soutien d'étiage. Ensuite, face à la multiplication des phénomènes violents et extrêmes, en montagne certainement plus qu'ailleurs, je vous rappelle l'impérieuse nécessité de préserver les stations locales de Météo France, comme celles de Chamonix, de Bourg-Saint-Maurice ou de Briançon, ... Très bien ! ... encore menacées à ce jour. Au-delà de leur fonction de prévision météo, ces antennes locales sont incarnées par des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire, de ses zones à risque, ainsi que de l'évolution des conditions nivologiques en période de crise. Elles fournissent, depuis des décennies et de manière irremplaçable, une prévision météo déterminante pour prévenir la survenance d'événements climatiques pouvant affecter la sécurité des populations. Dans ces circonstances, la délocalisation de ces trois antennes locales vers un centre grenoblois serait un non-sens qui affecterait gravement le niveau de prévision et, donc, l'adaptation des mesures

mais aussi des rôles d'aménagement du territoire et de gestion hydraulique. C'est bien la complexité de ces différentes fonctions que nous mettons en avant dans nos échanges en cours avec la en cours avec la Commission européenne sur le devenir de nos concessions hydroélectriques. C'est également ce que nous avions mis en avant dans les discussions qui ont été conduites sur la prolongation de la concession de la CNR. CNR. Je partage donc tout à fait votre avis sur l'importance de ces concessions d'hydroélectricité, dont le rôle va très au-delà de la simple production d'électricité, qui ne peut pas être appréhendée sous ce seul prisme. S'agissant de Météo France,

investissements. Ces nouveaux outils technologiques au service d'une meilleure prévision météo pour l'ensemble de nos concitoyens ont forcément des conséquences sur l'organisation de Météo France, en particulier sur son implantation territoriale. J'ai bien en tête la présence d'agents à Bourg-Saint-Maurice, à Chamonix ou à Briançon. Les réflexions sur la réorganisation de Météo France, Météo France, fondée sur des nouveaux outils, peuvent conduire à remettre en cause des implantations locales, mais le sujet des Alpes est pris très au au sérieux. Des échanges se tiendront dans les prochains jours avec la nouvelle présidente-directrice générale de Météo France et les élus afin de voir quelles solutions peuvent être trouvées pour les agents actuellement présents dans ces communes.

Stéphane Piednoir. Parmi les recommandations de l'excellent rapport de nos collègues, plusieurs d'entre elles convergent vers une nécessaire optimisation de la politique de rénovation thermique des logements et, plus globalement,

il faut clarifier le rôle des différentes structures et des différents acteurs dans le domaine et les accompagner. Or, aujourd'hui, les initiatives sont multiples et, en définitive, souvent illisibles, voire suspectes aux yeux du grand public. Vous l'avez vous-même évoqué, madame la ministre, c'est un véritable parcours du combattant. Comme vos collègues Emmanuelle Wargon et Julien Denormandie, que j'ai eu l'occasion d'interpeller à ce sujet lors d'un congrès à Angers, vous citez les régions et les intercommunalités pour assumer ce rôle de pilote sur des programmes d'actions concrètes,

L'idéal serait sans doute de couvrir l'ensemble du territoire de structures portées par les collectivités, à l'instar des ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat, et, surtout, dotées de moyens humains et financiers pérennes, qui ne seraient pas soumis aux fluctuations de financements de l'Ademe, avec la fixation d'objectifs réalistes. De manière complémentaire, cette ambition me semble devoir être partagée avec les professionnels de la construction, perdus, perdus, eux aussi, parmi les labels et autres normes qu'on leur propose ou impose trop souvent. Madame la ministre, quelle est votre vision territoriale de la décentralisation des politiques publiques dans le domaine de la rénovation thermique ? Merci de conclure, cher collègue ! Qu'en est-il du plan, annoncé par vos collègues, de rénovation des établissements scolaires, qui sont souvent de véritables passoires thermiques ?

de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela montre à quel point ce secteur joue un rôle crucial pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments publics doivent être

et des soutiens au travers de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Je fais le constat que, dans certains départements, les actions de rénovation énergétique des écoles ont été largement engagées. Tel n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on peut s'interroger sur la façon de donner une plus forte dynamique à ces actions de rénovation énergétique de nos bâtiments publics.

par une simplification des dispositifs d'aide. Je continue à penser que devoir conjuguer des aides de l'ANAH, un crédit d'impôt, des certificats d'économie d'énergie, des éco-PTZ

Ayons aussi à l'esprit que le climat est un sujet extrêmement complexe, qui appelle de nous des actes concrets, mais aussi beaucoup d'humilité. Le très bon rapport d'information de la délégation sénatoriale à la prospective aborde un sujet au coeur des tensions territoriales, déjà largement évoqué ce matin, l'adaptation des politiques de l'eau, sujet d'actualité après les deux canicules de l'été 2019 et la sécheresse qui a entraîné des mesures importantes de restriction d'eau dans nombre de nos territoires. Les politiques de l'eau doivent donner la priorité à des usages plus économes de la ressource et à la mise en oeuvre de solutions fondées sur la nature pour optimiser la la recharge des nappes phréatiques et développer des équipements hydro-économes. Quatre options permettent de mieux exploiter l'eau excédentaire des saisons pluvieuses : barrages-réservoirs, ouvrages en lit mineur, de type moulins, étangs ou plans d'eau, retenues collinaires, qui stockent le ruissellement, ruissellement, restauration de zones humides naturelles. Pourtant, aujourd'hui, en vertu d'un plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'administration de l'eau a détruit plus de 150 petits barrages sur nos rivières depuis dix ans. Les conséquences d'une telle décision sont nombreuses : assèchement de rivières, disparition ou réduction d'une grande partie de la faune piscicole, fragilisation de bâtis, baisse de la nappe alluviale et disparition de certaines zones humides, avec des modifications d'écosystèmes et de biodiversité dans les vallées ayant un impact sur l'agriculture et le tourisme. Madame la ministre, pour adapter la France aux dérèglements climatiques, nous devons nous appuyer sur le local, mais aussi sur ce patrimoine hydraulique. Quelle nouvelle politique de protection et de valorisation des ouvrages hydrauliques envisagez-vous ?

l'eau qui n'est pas retenue, par le biais de barrages de stockage ou de retenues collinaires, a un rôle très important pour alimenter nos nappes phréatiques, soutenir en aval les débits des cours d'eau

de tout faire pour améliorer les capacités d'infiltration, limiter le ruissellement, préserver nos milieux humides et restaurer les capacités d'écoulement de nos cours d'eau. Monsieur le sénateur, vous évoquez les politiques

de nos ouvrages hydrauliques qui stockent l'eau afin de recharger les sols et les nappes en eau, de recréer des milieux aquatiques et des zones humides qui contribuent à la production de biodiversité. En effet, la reconquête de la biodiversité terrestre et marine permet de lutter contre le dérèglement climatique. Pour

climatique, qui menace directement les activités au coeur de l'économie montagnarde que sont le pastoralisme et le tourisme. Madame la ministre, vous avez évoqué dans votre introduction les risques naturels en montagne. Il s'agit d'un sujet important ces risques vont s'accroître du fait du réchauffement climatique et il faut adapter les outils de prévention. L'impact du réchauffement climatique va bien au-delà du risque naturel. J'appelle l'attention sur le fait que le plan national d'adaptation au changement climatique doit créer les outils